qui témoigne d'abord d'une volonté forte, partagée au Sénat comme à l'Assemblée nationale, de faire aboutir cette réforme du système ferroviaire français, indispensable et très attendue. Ce texte comporte plusieurs avancées que nous soutenons : il pose les conditions de l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, il met fin au recrutement au statut de cheminot à compter du 1 janvier 2020 et il transforme les établissements publics qui composent le groupe public ferroviaire en sociétés anonymes. Cet accord témoigne aussi d'un échange fructueux entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je le rappelle, le projet de loi initial comportait huit articles, essentiellement des articles d'habilitation à procéder par ordonnances il en compte désormais trente-cinq, et les principales habilitations ont été remplacées, au cours de la navette, par des dispositions législatives modifiant directement le droit en vigueur. Au Sénat, nous avions adopté dès le départ une attitude constructive à propos de ce texte. Je veux d'ailleurs saluer la qualité du dialogue que nous avons pu avoir avec vous, madame la ministre, pour préciser les dispositions introduites à l'Assemblée nationale et les compléter, en particulier sur le volet social ; j'y reviendrai. Cette façon de travailler nous a permis de nous concentrer, en commission mixte paritaire, sur les quelques points de divergence subsistant entre les deux assemblées. Je veux à cet égard remercier le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Djebbari, avec qui nous avons beaucoup échangé pour préparer cette CMP. Je me réjouis d'autant plus de cette large majorité que le texte issu de la CMP préserve l'essentiel des apports du Sénat. Pour mémoire, nous avions enrichi ce texte selon quatre objectifs

maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté au sein du système ferroviaire. En matière d'aménagement du territoire, le texte issu de la CMP conserve l'obligation faite à l'État de conclure des contrats de service public pour préserver la desserte TGV des villes moyennes sans correspondance. Sur le volet social, la CMP a maintenu le cadre relatif au transfert des salariés vers de nouveaux opérateurs, auquel le Sénat avait apporté des compléments significatifs. Je le rappelle, le dispositif que nous avons adopté favorise le recours le plus large possible au volontariat des salariés pour rejoindre les nouveaux opérateurs et garantit aux salariés transférés le maintien de droits sociaux substantiels. En ce qui concerne l'effectivité de l'ouverture à la concurrence, le texte de la CMP conserve des apports majeurs du Sénat du Sénat : le rattachement de Gares & Connexions sous la forme d'une filiale de SNCF Réseau disposant d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière et qui contractualisera directement avec l'État sur des objectifs propres aux gares l'extension du champ des informations qui devront être transmises par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure et des gares aux autorités organisatrices de transport, sur le modèle de ce que prévoyait la proposition de loi du président Maurey et de notre ancien collègue Louis Nègre ; le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance aux autorités organisatrices de ; l'encadrement de deux dérogations trop générales à l'obligation de mise en concurrence des services conventionnés. Seuls trois sujets ont fait l'objet d'une évolution notable en commission mixte paritaire. concerne le transfert des salariés, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoyait que le nombre de salariés à transférer soit arrêté par l'opérateur sortant. Or il nous semblait important que les régions puissent avoir leur mot à dire et demander que ce nombre soit corrigé si elles estiment qu'il ne correspond pas aux besoins d'exploitation du service ferroviaire.

Le deuxième sujet concerne l'indépendance de SNCF Réseau. Pour que l'ouverture à la concurrence réussisse, il est nécessaire de garantir l'indépendance de SNCF Réseau, afin que l'ensemble des opérateurs aient un accès équitable aux infrastructures ferroviaires. Pour ce faire, le Sénat a renforcé le régime d'incompatibilité des fonctions de membre du conseil d'administration et de surveillance ou de dirigeant de SNCF Réseau avec l'exercice de telles fonctions au sein d'une entreprise ferroviaire. Étant donné que SNCF Réseau restera intégré, avec SNCF Mobilités, au sein d'un même groupe, il nous est apparu nécessaire que l'indépendance de SNCF Réseau soit également assurée à l'égard de la SNCF. Il serait en effet inconcevable que le président de SNCF Réseau puisse continuer d'exercer des missions dirigeantes au sein de la. En CMP, nous avons préservé cette indépendance du président et des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau à cet égard de la. étant donné que cette exercera pour le compte de SNCF Réseau certaines missions transversales, nous avons permis que certains dirigeants de SNCF, par exemple son directeur financier, puissent siéger au conseil d'administration de SNCF Réseau. Enfin, la CMP est parvenue à un équilibre sur la question de la tarification du réseau. Elle a supprimé l'avis conforme de l'ARAFER sur le volet tarification du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau que le Sénat avait introduit, mais elle a préservé un mécanisme incitatif pour éviter le blocage de la tarification du réseau en cas d'absence de validation de la tarification annuelle par l'ARAFER en temps utile. SNCF Réseau devra tout d'abord présenter un nouveau projet de tarification dans un délai de trois mois, pour que le régulateur puisse à nouveau se prononcer avant le début de l'horaire de service. En cas de persistance du désaccord, le texte issu des travaux du Sénat avait prévu la reconduction de la tarification antérieure sans indexation sur l'inflation. Pour éviter de trop mettre en difficulté SNCF Réseau, nous avons finalement accepté la reconduction de la tarification indexée sur l'inflation, mais pendant une année seulement. Si le désaccord devait persister pendant plusieurs années- ce que nous ne souhaitons bien évidemment pas -, la tarification serait gelée et ne pourrait plus être indexée les années suivantes. Cela incitera donc SNCF Réseau à fournir tous les efforts requis pour présenter une tarification conforme au droit européen, et par conséquent acceptable par l'ARAFER. Vous le voyez, mes chers collègues, l'essentiel des apports du Sénat sur ce texte a été conservé en CMP, en vue de permettre une ouverture à la concurrence ambitieuse, qui respecte les droits des salariés et qui maintient la desserte de nos territoires. Nous pouvons nous réjouir que la voix du Sénat ait été entendue sur ce texte et que cela ait permis d'enrichir cette réforme sur des points substantiels. Je forme le voeu, madame la ministre, que cette démarche d'ouverture du Gouvernement à l'égard de la Haute Assemblée se poursuive à l'avenir. ! Pour conclure, je veux encore une fois m'adresser solennellement aux grévistes. Désormais, la loi est votée, la grève ne sert plus à rien.

je ne citerai ni Victor Hugo, ni Jules Renard, ni Maurice Thorez, monsieur le rapporteur, mais Portalis, qui veille sur la qualité des travaux de la Haute Assemblée Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires. » Vous avez, nous avons, mesdames, messieurs les sénateurs, écrit une loi nécessaire : nécessaire pour nos concitoyens, qui attendent un meilleur service public ferroviaire, au meilleur coût nécessaire pour donner aux régions les leviers dont elles ont besoin pour mettre pleinement le train au service des territoires ; nécessaire pour conforter le statut public de la SNCF tout en lui donnant la souplesse d'une véritable entreprise, responsable de son destin ; nécessaire enfin pour garantir aux cheminots que l'ouverture à la concurrence s'accompagnera d'un cadre social protecteur. Depuis l'annonce du nouveau pacte ferroviaire, le 26 février dernier, j'ai mené cette réforme, tenu le cap avec détermination, dans un esprit de dialogue, fidèle à la méthode que le Premier ministre avait annoncée. La loi que vous vous apprêtez à voter repose sur des principes structurants. Le premier est l'ouverture à la concurrence. Cette concurrence, vous l'appeliez de vos voeux, conscients comme moi qu'elle n'est pas une menace pour la SNCF. Comme vous, j'ai confiance en la SNCF, que je sais forte de ses quatre-vingts ans d'histoire et capable des plus grandes prouesses. J'ai confiance dans les cheminots, ces 150 000 femmes et hommes dont je connais l'engagement au quotidien. Cette concurrence, vous l'avez voulue progressive dans son calendrier et protectrice, tant pour les salariés, en cas de changement d'opérateur, pour les territoires, en maintenant une desserte fine et pour les usagers, en restant intransigeant sur les impératifs de sécurité. Cette concurrence n'a qu'un but : donner à nos concitoyens accès à plus de trains et à des trains moins chers. Le second principe de cette réforme est la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics, pour en faire un groupe industriel performant et un champion sur ce marché. Détenue à 100 % par l'État, avec des capitaux incessibles, la SNCF est et restera publique. Il n'est pas responsable d'agiter des peurs quand, sur toutes les travées de la Haute Assemblée et sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, ce principe est unanimement partagé. C'est la plus sûre des garanties. Cette réforme permet également de refonder le pacte social des cheminots pour l'adapter, dans une logique d'équité, à un monde ouvert à la concurrence. En un mot, cette réforme pose les bases d'un système ferroviaire que nous souhaitons résolument tourné vers l'avenir et incarnant pleinement cette valeur fondamentale du service public qu'est l'adaptabilité aux besoins des territoires et des citoyens. Certains voudraient agiter des épouvantails, entretenir la confusion, pour mener des combats qui ne servent ni les cheminots ni le service public ferroviaire. Je le redis, le contrat moral passé entre la SNCF et les cheminots sera respecté, et des garanties de haut niveau sont apportées aux cheminots en cas de transfert. Enfin, le Gouvernement, prenant pleinement ses responsabilités, a présenté les leviers nécessaires pour redresser le modèle économique de la SNCF et lui donner tous les atouts pour s'engager résolument dans l'avenir. l'élaboration de cette réforme, fidèles à ces principes et à la méthode que nous avions annoncée afin de répondre à l'urgence de la situation. En effet, le Gouvernement a présenté un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnances. Dès l'examen du texte à l'Assemblée nationale, les principales modalités de la réforme ont pu être inscrites dans le texte ; vous les avez complétées et précisées, dans un travail inédit de coconstruction. Cette méthode, vous le savez, a permis de prendre pleinement en compte le fruit d'un dialogue structuré et permanent avec les organisations syndicales et les collectivités.

Vous l'avez fait en intégrant dans le texte, sans remettre en cause les principes de la réforme, les propositions issues de la concertation. Sans renier leur opposition aux fondamentaux de cette réforme, certains syndicats ont ainsi permis d'apporter aux cheminots des garanties concrètes

Mesdames, messieurs les sénateurs, le 5 juin dernier, vous avez refusé l'immobilisme dans lequel certains voudraient enfermer le service public ferroviaire et avez adopté un texte majeur. Cette réforme traduit un engagement sans précédent du Gouvernement en faveur du transport ferroviaire : engagement déterminé, avec le refus de la facilité d'une réforme engagement

Cet engagement ne s'arrêtera pas après le vote de ce matin. Il reste, vous le savez, au sein de la branche, un travail important à mener pour les partenaires sociaux, auxquels il revient de dessiner un cadre social commun et protecteur. Comme vous, j'en appelle à la responsabilité. La tâche est importante, le calendrier est ambitieux, mais réaliste. Je veux croire que les organisations syndicales et patronales seront à la hauteur des attentes des salariés du secteur. Je l'ai indiqué, il n'appartient pas à l'État de se substituer aux partenaires sociaux ; pour autant, je serai particulièrement vigilante au bon déroulement de la négociation, que je relancerai, demain après-midi, en réunissant organisations syndicales et patronales au ministère des transports. Par ailleurs, comme je m'y suis engagée, monsieur le rapporteur, vous serez étroitement associé au travail de rédaction des ordonnances techniques, pour lequel la Haute Assemblée va habiliter le Gouvernement. Enfin, je veillerai à ce que le rapport attendu sur les « petites lignes » ne vienne pas nourrir la longue liste des rapports non remis. Je m'y engage personnellement, car il sera un outil important pour le Gouvernement, le Parlement et les régions.

et le président de votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey. Nous avons travaillé dans un climat de confiance constructif. Cette confiance s'est traduite dans la qualité de nos débats, riches, passionnés mais respectueux. Ce climat a également prévalu, je le sais, dans vos échanges avec vos collègues députés issus de la majorité gouvernementale lors de la commission mixte paritaire, et je m'en félicite. Enfin, je veux de nouveau saluer devant vous l'attention particulière portée par le président Larcher à cette oeuvre commune. Mesdames, messieurs les sénateurs, Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est soumis est le résultat d'une ambition claire du Gouvernement, déterminé sur les principes d'une volonté partagée de donner toute leur place aux propositions des partenaires sociaux ouverts au dialogue, d'un enrichissement permis à chacune des étapes du débat parlementaire par un dialogue permanent et exigeant entre le Gouvernement et le Parlement. Le texte que vous vous apprêtez à voter est le premier volet d'un projet qui, vous le savez, me tient à coeur : le projet de loi d'orientation des mobilités. Je sais que celui-ci est attendu ; il traduira l'engagement du Président de la République en faveur d'une société de la mobilité ; je le présenterai cet été. Il contribuera, lui aussi, à répondre à la triple exigence que vous partagez : une exigence de justice pour nos territoires et nos concitoyens les plus fragiles une exigence d'efficacité, avec la loi de programmation qui traduira la priorité qui m'anime, celle d'améliorer la mobilité du quotidien une exigence environnementale, enfin, pour tenir nos engagements- je pense aux accords de Paris mais aussi à la santé et au bien-être de nos concitoyens. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il est des moments qui comptent plus que d'autres dans une vie de parlementaire, et l'élu que je suis, qui n'en est pas encore à une année pleine de mandat, mesure toute l'importance de cet instant. tout n'a pas été un long fleuve tranquille depuis le 26 février dernier, date à laquelle, madame la ministre, vous avez donné avec le Premier ministre le coup d'envoi de la réforme ferroviaire. Pour la première fois depuis bien des années, un gouvernement, celui que j'ai l'honneur de soutenir, décidait de mettre fin aux atermoiements, aux renoncements, et de s'attaquer frontalement à la réforme d'un système ferroviaire en bout de course. Oui, ce que vos prédécesseurs n'ont pas voulu faire, madame la ministre, vous avez eu l'audace et le courage de l'entreprendre, pour garantir un avenir au service public ferroviaire français face à l'ouverture à la concurrence. De l'audace, il fallait en avoir pour s'attaquer à un sommet aussi ardu que celui de la réforme du système ferroviaire. Du courage, il en fallait aussi pour bousculer ces habitudes et ces corporatismes qui caractérisent trop souvent notre système français. Je parle d'audace, je parle de courage ; j'y ajouterai la volonté farouche et permanente de trouver la solution législative la plus efficiente et la plus pertinente pour notre modèle français. Cette solution a été trouvée dans le cadre de ce travail de coconstruction entre le Gouvernement et nos deux assemblées, notamment le Sénat, qui a joué un rôle essentiel. C'est l'occasion pour moi de saluer une nouvelle fois le travail d'orfèvre réalisé par notre rapporteur Gérard Cornu sous la houlette bienveillante du président Hervé Maurey. Hervé Maurey. La commission mixte paritaire a permis de mesurer tout l'apport du travail sénatorial en s'accordant sur un texte parfaitement équilibré, qui fait la part belle à l'efficacité, à la modernité et à la justice sociale. justice sociale, oui, car la Haute Assemblée a fait la démonstration que « penser social » n'est pas que le drapeau de quelques-uns, qui en font l'alpha et l'oméga d'un logiciel politique qu'ils peinent d'ailleurs à réinventer. Nous avons montré notre attachement au monde cheminot au travers de dispositions fortes mettant en place des garanties sociales de haut niveau pour les cheminots qui seraient concernés par un transfert vers un nouvel opérateur. Nous avons noué avec les organisations syndicales réformistes un dialogue fécond qui a permis d'améliorer considérablement le texte, dans un travail de coconstruction de tous les instants. La transformation de la SNCF en un groupe unifié dont les capitaux seront intégralement détenus par l'État et incessibles garantit un service public ferroviaire moderne et plus performant, et permet de mettre un terme à toutes les polémiques. L'unité sociale de ce groupe unifié est affirmée, répond aux attentes des organisations syndicales, et chacun se félicitera que ce soit au Sénat que cela a été précisé. Non, l'ouverture à la concurrence n'est pas une fatalité pour notre service public ferroviaire

pour la desserte des territoires et garantissent la défense des intérêts des usagers, avec notamment l'institution de comités de suivi des dessertes auprès des autorités organisatrices de transport. L'efficacité, c'est aussi le renforcement de la règle d'or, à la suite de l'annonce de la reprise progressive de la dette. Accompagnée d'un engagement fort de l'État dans le domaine de l'investissement, elle doit contribuer à sécuriser la trajectoire financière de la SNCF, et chacun ici ne pourra que s'en féliciter. N'en déplaise à certains, le Gouvernement a pris toutes ses responsabilités en matière financière pour permettre à cette octogénaire respectable et respectée qu'est la SNCF d'appréhender l'avenir. Tous les ingrédients sont désormais réunis pour permettre une ouverture à la concurrence qui sera profitable à tous et pour permettre à notre société nationale d'écrire une nouvelle page de son histoire, de notre histoire.

Il en est ainsi du devenir des gares dans le domaine des intermodalités et d'un futur qui se doit d'être radieux. La gestion plus efficace des gares, avec la mise en place d'une filiale de SNCF Réseau, doit permettre de conforter le rôle de ces places fortes de notre système ferroviaire et d'en faire des lieux de vie incontournables dans notre paysage quotidien. La gare est un élément essentiel de l'aménagement du territoire et la coconstruction de son avenir avec celles et ceux qui vivent autour d'elle est une condition primordiale de la réussite des mobilités de demain. « Peut-être le bonheur n'est-il que dans les gares ? », disait Georges Perec. Voilà en tout cas un sujet sur lequel nous avons moult propositions à formuler. Nous aurons aussi à reprendre le sujet de la distribution des titres de transport et à nous pencher sur celui de la numérisation, en nous inspirant sans doute d'exemples européens. Cette réforme ferroviaire est l'acte I du grand chantier des mobilités, et nous en avons fait un atout pour les débats à venir. Le nouveau pacte ferroviaire que nous allons adopter apporte, je le disais, des garanties fortes aux cheminots, dont on peut bien évidemment comprendre et partager les interrogations, tout à fait légitimes. Le Gouvernement a donné par votre intermédiaire, madame la ministre, des garanties complémentaires quant aux négociations entamées dans le cadre de l'élaboration de la convention collective de la branche ferroviaire et quant au rôle que l'État entend tenir dans ces négociations. Le moment est donc venu, Gérard Cornu le disait, de mettre un terme à une situation qui paralyse l'économie du pays et handicape considérablement celles et ceux de nos concitoyens pour qui le train est le seul moyen de se rendre sur leur lieu de travail.

Loin de moi l'idée de faire tel ou tel procès d'intention, ... C'est raté ! ... mais cette situation n'a que trop duré, car elle fragilise davantage encore notre société nationale et celles et ceux qui en sont les acteurs, les cheminots. Nous devrions au contraire nous satisfaire que la représentation nationale ait pleinement joué son rôle pour mettre au point un texte qui grave dans le marbre notre attachement indéfectible au service public ferroviaire. Bien évidemment, le groupe La République En Marche votera ce texte. La

Si nous pouvons avoir des divergences d'opinions, nous devons respecter le cadre démocratique de nos débats et accepter la confrontation d'idées, sans qu'elle donne lieu à des insultes. Ces paroles et ces actes n'honorent pas ceux qui s'y prêtent dans cette enceinte républicaine. Cette mise revenons-en à ce qui nous occupe ce matin : la clôture des débats parlementaires sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Cette clôture est toute provisoire, puisqu'il nous faudra ratifier l'ensemble des nombreuses ordonnances prévues par le présent texte lors de la prochaine session parlementaire. À cette occasion, je vous le dis,

Ce n'est pas une surprise : tout au long des débats, nous avons constaté une volonté commune à la majorité présidentielle et à la majorité sénatoriale d'en finir avec la culture publique du rail dans notre pays en changeant le statut de l'opérateur national, la SNCF, et en libéralisant la quasi-totalité des transports de voyageurs. Nous le regrettons, pour les territoires comme pour les usagers du rail, car, au-delà des discours, la libéralisation s'accompagne toujours d'une dégradation du service, de l'abandon des activités non rentables, d'un changement de logique. Je n'en prendrai qu'un exemple, celui du gaz, particulièrement éclairant, si je puis dire

pour les années 2009 à 2016. Cela fait beaucoup de pognon, comme dirait l'autre ... Dans le même temps, le taux de participation des salariés était de 1 %. Quant aux tarifs, ils ont augmenté de 80 %. Nous ne voulons

Les cheminots restent, avec lucidité et dans l'unité de leurs forces syndicales, extrêmement mobilisés pour refuser ce nouveau pacte ferroviaire. Les pseudo-garanties apportées, notamment en cas de transfert, n'auront donc pas suffi à rassurer les agents du service public. Les amendements « très sociaux », comme les qualifiait le rapporteur, n'auront pas pu cacher le sombre dessein qui sous-tend ce projet de loi : la fin programmée du statut et le renvoi à une nouvelle convention collective, dont il n'est absolument pas évident qu'elle soit aussi favorable aux salariés.

c'est la fin des cars Macron. En contradiction avec ses engagements européens et internationaux, la France n'a pas respecté la trajectoire fixée pour ses émissions de gaz à effet de serre, notamment pour ce qui concerne les transports. C'est incompréhensible. L'avenir, ce sont des trains plus nombreux, notamment des trains d'équilibre du territoire, pour lutter contre l'enclavement et la désertification rurale. L'avenir, ce sont des trains plus sûrs et plus ponctuels. En effet, mes chers collègues, il ne faut pas imaginer une seule seconde que cette réforme va changer quoi que ce soit à la galère quotidienne des usagers. Moderniser le service, c'est moderniser le réseau et les installations, aujourd'hui vétustes et obsolètes, ... Là, nous sommes les chutes de caténaire, les pannes, à l'instar de celle qui, hier encore, est survenue à Saint-Lazare. À cela, la concurrence ne changera rien. Ce qu'il faut, ce sont donc des financements. À cet égard, les sommes annoncées par le Gouvernement ne sont que de simples promesses, notamment pour ce qui concerne l'avenir des lignes de vie dans le cadre des contrats de plan.

l'État de près de 2 milliards d'euros de ressources, qui vont dans la poche des actionnaires. Vous n'avez pas voulu vous saisir de ces outils, préférant renvoyer ces questions à plus tard. Alors, nous prenons date, et nous reformulerons toutes ces propositions d'avenir lors de l'examen du projet de loi

un excellent travail sur ce texte, les membres de la commission mixte paritaire et, d'une façon générale, tous les acteurs qui ont contribué à l'aboutissement de ce dossier réellement difficile. Le « pacte ferroviaire » figurera sans doute parmi les textes les plus importants du quinquennat. Qu'on le soutienne ou qu'on le combatte, son adoption laissera des traces, et l'on s'en souviendra. Cela ne surprendra personne, les élus du groupe Union Centriste, au nom duquel je m'exprime aujourd'hui, font partie de ses soutiens-

Un consensus pourrait-il enfin se dégager sur cette réforme si clivante ? Force est de constater, à l'issue de la discussion parlementaire de la réforme, que le débat n'a pas été confisqué par le Gouvernement. À l'origine, nous avions pourtant de bonnes raisons de le craindre. La décision de l'exécutif de sortir la question ferroviaire du champ du projet de loi-cadre sur les mobilités et de la traiter par voie d'ordonnances, alors même que le Sénat, sous la houlette d'Hervé Maurey et de Louis Nègre, avait déjà beaucoup travaillé sur le sujet, n'était pas de très bon augure. Mais nous avons été entendus. Le texte a été débattu, travaillé, il a cheminé. Chacun a pu exprimer sa sensibilité et ses convictions : le débat parlementaire a bien eu lieu. Nous vous en remercions une nouvelle fois, madame la ministre. Le champ des ordonnances s'est finalement restreint aux questions les plus techniques, ce qui correspond à leur raison d'être. Le législateur a pu jouer son rôle en précisant les grandes lignes de l'ouverture à la concurrence, du statut des salariés et de la prise en compte de l'aménagement du territoire. Le Sénat, en particulier, a pesé de tout son poids dans la discussion. L'historique de cette réforme prouve une fois de plus, s'il en était besoin, l'utilité fondamentale, pour la démocratie, de la chambre haute et de ses apports. Je n'ai pas d'observations particulières à formuler sur les trois points qui restaient à trancher en commission mixte paritaire. Nous sommes favorables aux derniers aménagements apportés en termes de gouvernance des trois sociétés. Nous nous réjouissons que les pouvoirs de l'ARAFER en matière de tarification du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau aient été préservés. Enfin, concernant la fixation du nombre de salariés à transférer en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public, sujet qui avait suscité de vifs débats en commission et en séance, il ne nous paraissait pas très rationnel que cette tâche importante incombe au seul opérateur historique. Quand on perd un marché, on n'impose pas ses conditions au nouvel entrant C'est pourquoi le en vertu duquel le nombre de salariés à transférer en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public sera déterminé d'un commun accord par l'autorité organisatrice et par l'opérateur sortant nous convient beaucoup mieux, d'autant que cette démarche est par nature tout à fait centriste

qui ne sont pas des moindres : inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans les objectifs de la SNCF ; garantie de l'unité sociale par la création d'un même socle de droits au sein de l'ensemble du groupe ; extension de six à huit ans du délai durant lequel les salariés transférés aux nouveaux opérateurs pourront pourront demander à réintégrer le statut en cas de réembauche au sein du groupe SNCF. Ce sont là des mesures qui devraient contribuer à éteindre l'incendie social et à rassurer les plus inquiets. Mais, parce que le temps législatif n'est pas toujours celui de l'acceptation sociale, nous sommes bien conscients, madame la ministre, qu'il vous faudra encore faire preuve de beaucoup de pédagogie. Une fois les écritures couchées sur le papier, il faut encore évangéliser Le Sénat a aussi apporté sa pierre sur des sujets plus techniques et pratiques, de la plus grande importance : le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance, la vente des billets, le maintien d'un haut niveau de sécurité et de sûreté. j'ai gardé pour la fin le volet qui me tient le plus à coeur, et qui retient toute l'attention des représentants des territoires que nous sommes : celui de la desserte des zones rurales et de l'avenir de ce que l'on appelle « les petites lignes », au-delà des incertitudes qui pèsent sur certaines lignes TGV. Je vous avoue avoir participé à nos discussions sans perdre de vue le risque qu'une telle réforme pouvait présenter pour la vitalité de nos territoires. L'ouverture à la concurrence, oui, mais pas à n'importe quel prix ni à n'importe quelles conditions. Il faut savoir que, quand une zone rurale perd son train, sans disposer d'une solution de rechange, elle sombre dans l'enclavement. Or l'enclavement- chacun en a bien conscience dans cet hémicycle -a des conséquences lourdes, rapides et irréversibles. Les offres de mobilité peuvent et doivent être diverses et complémentaires, nous le savons. Mais, dans un contexte où l'avenir des lignes secondaires est incertain, l'entretien des routes problématique, les déplacements en voiture toujours plus lents et plus chers, les investissements verrouillés par des logiques comptables, les ruraux doutent désormais de tout. Comment croire que des usagers moins nombreux auront droit à la même offre, ou en tout cas à une offre adaptée et suffisante ? Ces préoccupations ont été prises en compte dans le texte. Le Sénat a fermement réaffirmé le rôle de l'État pour préserver les dessertes d'aménagement du territoire. Ainsi, l'État pourra conclure des contrats de service public destinés à préserver à préserver les dessertes directes sans correspondance, même pour les lignes à grande vitesse. Il s'agit de garantir que l'ouverture à la concurrence dite « en » ne conduise pas à l'abandon pur et simple des dessertes moins rentables. De plus, les régions pourront contractualiser directement avec l'État et les opérateurs pour préserver les petites lignes. Enfin, le système de tarification est aussi conçu pour assurer une forme de péréquation entre les lignes les plus exploitées et celles qui le seront moins. Ces garde-fous étaient indispensables. Ils sont désormais en place. Seront-ils suffisants ? Ce n'est pas certain. C'est pourquoi, à titre personnel, je m'étais abstenue sur ce texte en première lecture. Le groupe Union Centriste, quant à lui, a fait le pari pascalien d'y croire, mais croyance ne rime pas avec blanc-seing. Nous ne continuerons de croire que ce que nous verrons. Maintenant que le temps législatif s'achève, s'annonce celui de la mise en oeuvre de la réforme dans nos territoires. Si nous sommes favorables à l'ouverture à la concurrence et si nous en attendons beaucoup,

depuis le début de nos débats, nous plaidons pour le fret ferroviaire : c'est le même réseau qui le porte et qui peut l'amortir. Il ne peut y avoir de nouveau pacte ferroviaire sans que cette question

d'autres monopoles, celui-ci estimant que « l'État n'a pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles ». Nous demeurons inquiets, et pour le moins perplexes.

Vous avez annoncé une reprise de la dette : très bien. Merci au gouvernement précédent de vous avoir permis de le faire, en ramenant le déficit de 5,2 % en 2012 à moins de 3 % en 2017

statut, la tête des cheminots. Quelle méthode, quel gâchis ! Pourquoi avoir ainsi brutalisé les cheminots et déclenché l'une des plus grandes grèves de la SNCF, qui n'est pas finie que de temps perdu ! Vous le savez, nous sommes favorables à l'ouverture maîtrisée à la concurrence. À ce titre, nous avions engagé d'importantes réformes en 2014 et voté le quatrième paquet ferroviaire en 2016. Les négociations sur la nouvelle convention collective du ferroviaire avaient été lancées en 2014.

On comprend leur anxiété, pour peu qu'on veuille bien la comprendre ! Nous aurions pu limiter encore, par le débat, le champ de cette cinquième ordonnance relative au transfert de personnels et au flou persistant.

Ce projet de loi n'est donc en rien la révolution ferroviaire annoncée. Premièrement, nous n'avons à ce jour pas de visibilité financière sur un nouveau modèle industriel et pérenne de relance du ferroviaire. Deuxièmement, rien n'est dit du fret. Troisièmement,

le champ social, avec la suppression brutale du statut des cheminots. Il y a confusion des genres. Ce nouveau pacte ferroviaire est aussi un nouveau pacte Les Républicains -En Marche, conclu sur le dos des cheminots. Madame la ministre, mes chers collègues, nous voterons contre les et nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines étapes : on ne gouverne pas la France comme on dirige une start-up !

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

Le projet de loi que nous étudions aujourd'hui est, par deux aspects, décisif pour l'avenir de ce pays. En premier lieu, il trace la route de l'avenir ferroviaire français en programmant l'ouverture à la concurrence et en en fixant les modalités pratiques.

Le texte issu de la commission mixte paritaire est le fruit de trois négociations menées avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Premièrement, il prévoit que le nombre de salariés à transférer en cas de changement d'attributaire d'un contrat devra être déterminé d'un commun accord. C'est une mesure qui satisfera les nouveaux entrants sur le marché, mais il faudra que l'ARAFER que l'ARAFER prenne toute la mesure de son rôle de garant de ces accords, pour que les employés du rail ne soient jamais lésés. Deuxièmement,

ne peut se faire qu'en accord avec une politique globale de développement durable et de préservation de l'environnement. Ce point est essentiel.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que nous abordons la dernière étape de nos débats sur la réforme du système ferroviaire, permettez-moi de revenir quelques instants sur la genèse Adopté par le Parlement européen en décembre 2016, le quatrième paquet ferroviaire prévoit l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs en Europe.

Des inquiétudes légitimes ont pu apparaître : il est question de libéraliser un service public, de transformer une entreprise nationale et de modifier les conditions de recrutement et de travail de ses agents. Les Français sont attachés à la SNCF et au service rendu chaque jour par les quelque 150 000 cheminots. Ils ont raison. Profondément européen, le groupe du RDSE s'est toujours montré, dans sa grande majorité, favorable à cette ouverture à la concurrence, aujourd'hui inéluctable et souhaitée par la plupart de nos concitoyens. Les conséquences en sont pour l'heure inconnues ; c'est la raison pour laquelle nous devons rester vigilants. Mais les défaillances du système actuel appellent une refonte en profondeur du rail français pour préserver son attractivité face aux autres modes de transport. Il s'agit d'un enjeu crucial en termes à la fois d'aménagement du territoire et de respect de l'environnement. Je ne reviendrai pas en détail sur les enjeux de ce projet de loi ; nous avons eu de nombreuses occasions d'en débattre. J'aurais souhaité davantage de garanties s'agissant des petites lignes qui maillent notre territoire. Il appartiendra aux autorités organisatrices, avec les moyens dont elles pourront disposer,

notamment en inscrivant dans la loi le caractère incessible du capital de la nouvelle société nationale SNCF. Cette précision aura le mérite de mettre fin à certaines rumeurs de privatisation imminente. qui est de la question du transfert des salariés de la SNCF vers un nouvel opérateur en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public, le Sénat avait apporté des garanties sociales, en concertation avec les syndicats.

Je note néanmoins avec satisfaction la volonté du Gouvernement et du Parlement de favoriser le plus possible le volontariat en cas de transfert. D'autres points ont fait l'objet d'une modification en commission mixte paritaire. Le nombre de salariés à transférer sera déterminé d'un commun accord par l'autorité organisatrice et l'opérateur sortant, avec possibilité de saisine de l'ARAFER en cas de différend. Ce compromis semble convenir au plus grand nombre.

La commission mixte paritaire a conservé en grande majorité les dispositions du texte issu des travaux du Sénat, lequel a pu, cette fois, prendre toute sa place dans le travail législatif. hérité d'un texte non abouti, mêlant habilitations à légiférer par ordonnances et dispositions modifiant directement le droit en vigueur, les sénateurs ont fait le choix de la transparence, en instaurant, au bénéfice des salariés, des collectivités et des usagers, des garanties fermes sur de nombreux plans. Le Gouvernement, de son côté, s'est montré inflexible sur les grands principes de cette réforme, mais a su apporter certaines clarifications, voire accepter certaines avancées, au gré des concertations qu'il a menées et du travail parlementaire. L'annonce de la reprise partielle de la dette et le retour à des investissements massifs dans la maintenance me semblent des pas importants pour l'avenir du ferroviaire : c'est sur ces points que doivent désormais se concentrer nos efforts. Le groupe du RDSE, satisfait d'avoir pu enrichir le projet de loi de certains de ses amendements, votera en grande majorité en faveur de l'adoption du texte. Toutefois, il restera vigilant quant au contenu des décrets à venir et au rôle joué par l'État dans les négociations de branche qui s'annoncent. Les rencontres tripartites qui débutent seront l'occasion, pour le Gouvernement, d'agir en faveur de l'instauration d'un socle commun de droits pour tous les salariés du nouveau système ferroviaire français. C'est en tout cas le souhait du groupe du RDSE. La parole

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, nous approchons du terme de nos débats sur un texte qui doit être le socle d'un nouveau pacte ferroviaire, le départ d'une réforme du groupe SNCF, à l'aube de l'ouverture du secteur du transport de voyageurs à la concurrence. Nous sommes extrêmement satisfaits que l'Assemblée nationale et le Sénat soient parvenus à un accord en commission mixte paritaire. Permettez-moi de vous dire ma satisfaction, en tant que membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, membre suppléant de la commission mixte paritaire, mais également petit-fils de cheminot. N'en déplaise à Mme Duflot, on peut être descendant de cheminot- cégétiste de surcroît -et considérer que, à un certain moment, il faut savoir terminer une grève,

grandeur nature : le Parlement est capable, sans contrainte, sans empêcher le Gouvernement d'agir, de voter dans les temps requis une réforme importante pour une entreprise nationale, son personnel et l'ensemble de nos concitoyens.

Le Sénat n'est pas aussi inutile que certains de vos amis se plaisent à le dire et à l'écrire ... Ça, c'est juste ! Cette loi donnera au Gouvernement les moyens d'agir pour d'agir pour ouvrir à la concurrence les services nationaux de transport de voyageurs dans le respect des directives européennes, d'une part, et pour adapter le groupe public SNCF à cette nouvelle donne, Avec ce texte, le Parlement donne au Gouvernement une base juridique, financière et comptable nouvelle qui doit permettre à la SNCF de s'adapter à l'ouverture du secteur à la concurrence, de montrer toutes ses capacités d'adaptation et de révéler son potentiel de productivité, qui lui permettra de rester une entreprise compétitive. Conscients des enjeux et misant sur la réussite de l'entreprise et de son personnel, nous avons d'ailleurs adopté le calendrier le plus souple possible. Il devrait permettre au groupe SNCF de relever ce défi. C'est une première étape, mes chers collègues, car il reste au Gouvernement à résoudre plusieurs questions déterminantes pour l'avenir du groupe SNCF et la garantie d'une véritable ouverture à la concurrence.

le Gouvernement s'est engagé à ce que l'État reprenne 35 milliards d'euros de dette de la SNCF. Même si, d'un point de vue comptable, il finira sans doute par obtenir que cette reprise de dette ne soit pas prise en compte pour le calcul du déficit public de la France, il n'en reste pas moins que le contribuable français devra payer, ainsi que les régions, selon toute vraisemblance. C'est la raison pour laquelle nous aimerions avoir des précisions sur les conditions de la reprise de dette en deux étapes et son « alignement » sur la productivité de l'entreprise. Deuxièmement, le changement de statut et la transformation de SNCF Mobilités en société anonyme ne doivent pas nous tromper : cette transformation restera accessoire si elle ne s'accompagne pas d'une réforme de structure et de management pour combler le déficit annuel d'exploitation, puisque la SNCF ne pourra plus bénéficier ni de la garantie implicite de l'État ni de sa notation en matière de dette. Il s'agit d'un vrai défi pour l'entreprise : être compétitive et se développer en réduisant son déficit d'exploitation, qui était de 2,5 milliards d'euros par an ces dernières années.

Cela vaut pour les prochaines négociations collectives de la branche ferroviaire et pour la réforme du régime de retraites que le Gouvernement promet d'intégrer dans la réforme globale à venir de notre système de retraites. Sur ces deux sujets, les enjeux sont réels. Le point d'aboutissement déterminera des règles, équitables ou pas, pour l'ouverture à la concurrence. Enfin, en tant qu'élu francilien, je ne peux m'empêcher d'évoquer la question du service minimum, notamment sur le réseau d'Île-de-France. dommage que le texte n'évoque pas cette question. Les utilisateurs des transports au quotidien y auraient été sensibles. Ce texte, loin de marquer un aboutissement, n'est donc qu'un point de départ pour la SNCF et l'avenir du ferroviaire dans notre pays. En conclusion, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

fait le choix de la responsabilité, afin que ce texte puisse être élaboré dans de bonnes conditions. Je crois, madame la ministre, que vous avez pu mesurer l'importance d'un dialogue bicaméral équilibré. J'espère que cette pratique inspirera vos collègues et que cette manière de travailler

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.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

Mme la ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous venez donc d'adopter à une très large majorité le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

à rénover en profondeur notre système ferroviaire pour apporter un meilleur service aux Français et à renforcer la SNCF, par un engagement sans précédent en termes d'investissements.

et de la délégation aux entreprises, de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, présentée par MM. Rémy Pointereau, Martial Bourquin et plusieurs de leurs collègues

M. le rapporteur a pris en compte, à juste titre, les petites communes, celles de moins de 10 000 habitants, mais en créant des strates de population avec plusieurs seuils pour étendre ces périmètres.

Les territoires ruraux ne sont pas systématiquement confrontés à la problématique du centre et de la périphérie. Les petites communes rurales peuvent fonctionner en réseau pour animer un territoire rural. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'instaurer un régime spécifique pour toutes les petites communes rurales, afin qu'elles puissent bénéficier du dispositif OSER, notamment lorsqu'elles se regroupent pour porter un projet commun de revitalisation. Dans ce cas, nous proposons que le projet soit porté par l'EPCI,

Qu'il y ait des initiatives gouvernementales, c'est très bien, mais nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte, en tant que tel, ce texte issu de travaux du Sénat.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, chers collègues, cet article vise, d'une part, à créer une agence dédiée aux centres-villes et centres-bourgs, dotée du statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial, et, d'autre part, à étendre la compétence de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, l'EPARECA, aux périmètres des opérations de sauvegarde et de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Je considère, à titre personnel, que cet article est d'une importance considérable relativement au sujet de la En effet, il semble que l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, l'ANCT, « mobilisera et coordonnera les moyens en ingénierie et en financements au profit des collectivités bénéficiaires Elle « aura vocation à donner davantage de lisibilité et d'efficacité à l'intervention de l'État dans les territoires » et permettra d'accompagner « en priorité dans leur démarche de réflexion stratégique et de montage de projet les territoires les plus en difficulté Or, à l'heure actuelle, nous sommes très éloignés d'une finalisation de la mise en place de cette agence, la lettre de mission indiquant que l'ANCT devra être opérationnelle, « au moins dans une première phase, à l'été 2018

l'extension de la compétence de l'EPARECA aux centres-villes faisant l'objet d'une convention « OSER » ne peut qu'être bénéfique pour les territoires, dans la mesure où cela implique un renforcement certain de ses effectifs et, surtout, de ses moyens. Il convient de rappeler que l'EPARECA n'a aucun projet en cours ni à venir sur le territoire martiniquais, et plus globalement dans les outre-mer, en dépit des programmes de rénovation urbaine menés notamment à Fort-de-France.

de l'EPARECA depuis 2016. C'était l'une des recommandations du schéma directeur d'urbanisme commercial qu'elle a réalisé et qui a été validé par toutes les collectivités locales partenaires.

les frais et qui rendent difficiles son action dans les centres-villes. L'EPARECA dispose d'un budget annuel de seulement 30 millions d'euros, dont une subvention de l'État s'élevant à l'insuffisante somme de 5,7 millions d'euros.

Pour la commission des affaires économiques, l'objectif essentiel est de soutenir l'ingénierie des territoires qui en ont le plus besoin. Pour atteindre cet objectif, on peut envisager plusieurs modalités d'organisation. Les auteurs de défendent l'idée que la revitalisation des centres-villes n'est qu'une composante de la cohésion des territoires. Nous sommes tout à fait d'accord sur le principe. le texte de la commission préfigure de façon assez méticuleuse la création d'une agence à l'action ciblée sur les centres-villes qui ont vocation à s'intégrer dans un ensemble plus vaste.

que nous examinons des grands chantiers lancés par le Gouvernement. Une préfiguration de l'agence nationale de la cohésion des territoires

de créer ces contrats de manière purement consensuelle. Le premier de ces outils, dénommé « bail à réhabilitation avec option d'achat

à loyer, mais à versement d'un montant forfaitaire, évidemment très faible au regard de l'état du logement. Afin que le preneur ne se trouve pas prisonnier d'un logement

Il s'agit tout d'abord de permettre à des personnes de s'installer dans un logement ancien nécessitant des travaux qu'elles s'engageraient à réaliser en échange d'un loyer réduit. d'un certain nombre de remarques sur les difficultés que pose le dispositif en matière de sécurisation juridique de l'opération et du preneur.

Cela passe par la rénovation de bâtiments anciens, de logements construits il y a plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Or ces rénovations sont très coûteuses.

chers collègues, si nous n'amenons pas des habitants dans les centres-villes et les centres-bourgs, tout ce que nous faisons ici ne servira à rien

S'agissant du 1° et du 3°, les auteurs de l'amendement reprenaient des dispositions, rejetées lors de l'examen en commission, qui appliquaient un taux réduit de TVA aux travaux réalisés dans le parc des logements privés, même lorsque ces travaux conduisent à rendre l'immeuble comme neuf.

partiellement social, la modification va dans le sens de ce qui avait été demandé par la commission. Elle nous paraît donc acceptable, puisque ne sont plus visés que le logement social et le logement intermédiaire, et non le logement privé.

Si l'on ne repeuple pas les centres-villes, tout ce que nous faisons ici sera voué à l'échec. Nous devons